mes chers collègues,

Parfois, les jeunes découvrent l’apprentissage un peu par hasard. Il faut en faire un choix d’ambition valorisé dans nos établissements scolaires, notamment dans nos collèges. Deuxième enjeu : l’adaptation des compétences. Les besoins des entreprises évoluent rapidement. Les transitions numérique, écologique, technologique et industrielle transforment les métiers et les attentes des entreprises. L’apprentissage, par sa souplesse et sa proximité avec le terrain, constitue l’une des meilleures réponses à ces mutations. et dernier enjeu : l’égalité des chances. L’apprentissage répond à un objectif de justice sociale ; chaque jeune, quels que soient son parcours, son lieu de vie, son origine, doit pouvoir accéder à un contrat, à un accompagnement de qualité, à un avenir professionnel vingtième édition des rencontres sénatoriales de l’apprentissage nous rassemble ce matin autour d’une conviction forte et partagée : l’apprentissage est une voie C’est une passerelle indispensable entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise. Plus encore, c’est un levier essentiel pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux de notre pays, aujourd’hui et à Je veux dire ici, devant les apprentis présents en tribune, qu’ils sont la preuve vivante que le talent n’a pas d’âge, que la détermination vaut tous les diplômes et que l’alternance entre l’école et l’entreprise forge des professionnels complets, complets, adaptables et responsables. En cela, les apprentis font la fierté de notre pays. Débattre des enjeux de l’apprentissage

nous soutenons tous l’apprentissage, qui est une chance, une ardente nécessité, une voie d’excellence, d’émancipation par le travail et de progrès pour nos sociétés et

La réforme issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a donc été couronnée d’un succès quantitatif indéniable. Le nombre important

France Compétences, chargée d’assurer la répartition et le versement des fonds, a constamment été en déficit depuis 2020. Le dernier budget de l’opérateur, adopté pour 2025, fait encore état d’un solde déficitaire d’un demi milliard d’euros. La commission des affaires sociales a pourtant été force de proposition pour assurer un équilibre financier à l’apprentissage, en suggérant de recentrer les dépenses de France Compétences sur ses missions premières. Le montant total des dépenses nationales en faveur de l’apprentissage est du reste devenu considérable, voire déraisonnable. En cumulant les dépenses de tous les financeurs, notamment des opérateurs de compétences, l’État et les régions, il atteignait 15,3 milliards d’euros en 2023. La rationalisation qui doit être opérée a déjà été engagée, mais elle doit être menée sans sacrifier la dynamique de l’apprentissage et sans mettre en difficulté les secteurs dans lesquels cette voie est une filière historique de formation.

l’idée de moduler les aides selon le niveau de qualification des formations suivies ne doit pas être abandonnée. La création de l’aide exceptionnelle lors de la crise sanitaire est allée de pair avec un soutien uniforme, quel que soit le niveau de formation.

qu’à ceux qui participent à leur formation. L’apprentissage est une expérience, tout le reste n’est qu’information, disait Albert Einstein. En France, l’apprentissage est une expérience ouverte aux jeunes de 16 à 29 ans, qui ont ainsi la possibilité de se former en alternance et de découvrir le monde du travail tout en préparant un diplôme reconnu par l’État.

des dernières années, les gouvernements ont développé l’apprentissage en accumulant les aides financières aux entreprises. Nous ne sommes évidemment pas opposés aux aides publiques à l’apprentissage, à condition que l’utilisation de ces aides Celles ci doivent servir à accompagner, à former le jeune à son futur métier. Selon l’économiste Bruno Coquet, les aides publiques à l’apprentissage étaient estimées à 25 milliards d’euros en 2023. d’euros en 2023. En trois ans, les entreprises ont, hélas ! vu les aides financières à l’apprentissage être divisées par quatre. En 2022, les entreprises recevaient 8 000 euros par apprenti. Depuis le mois de février dernier, la prime a été réduite à 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Je pense notamment, pour n’en citer que quelques uns, aux boulangers, aux bouchers, aux coiffeurs, aux ébénistes, aux métiers du commerce, de la restauration, de la communication ou du

L’apprentissage est plus qu’un dispositif de formation : c’est un levier stratégique pour répondre aux défis économiques, sociaux, écologiques et territoriaux qui sont devant nous. Il l’est pour les jeunes, pour les entreprises, pour les organisations et pour les territoires. Il l’est aussi pour la cohésion sociale et la souveraineté économique de notre pays. Je tiens à saluer la présence dans

Leur présence nous rappelle que, derrière les chiffres, il y a des visages, des parcours et des projets d’avenir. L’artisanat est un pilier essentiel de nos économies régionales comme de notre économie nationale. Il incarne à la fois la vitalité entrepreneuriale, la richesse de nos savoir faire et l’enjeu crucial de la transmission. En 2023, près de 20 % des apprentis des Pays de la Loire évoluaient dans le secteur artisanal. Ce chiffre illustre l’attractivité de ces métiers et nous appelle à penser un accompagnement à la hauteur derrière chaque maître d’apprentissage, il y a un engagement fort : former, transmettre, maintenir et développer des compétences. Cet engagement doit être reconnu, valorisé et soutenu. Cela implique une prise en

une politique de mobilité ambitieuse, car l’accès à un contrat d’apprentissage ne doit pas être conditionné à un lieu de résidence ou à des réseaux familiaux. Nous devons aussi élargir et adapter l’offre de formation, en lien avec les besoins des filières en tension. Je pense ici aux métiers des secteurs de l’animation, du social, des aides à domicile, dans lesquels la crise des vocations est profonde.

l’apprentissage doit être développé et reconnu. Cela suppose une concertation renforcée entre l’État, les régions, les branches professionnelles et les territoires. L’apprentissage demeure trop genré. Les filières industrielles ou artisanales demeurent majoritairement masculines, tandis que les secteurs du soin ou de l’éducation sont majoritairement féminins. Nous devons renforcer la féminisation de l’apprentissage et la mixité au sein de chaque filière, en luttant contre les stéréotypes, en améliorant les conditions d’accueil, en assurant la mixité dès l’orientation et en modifiant les représentations. L’essor de l’apprentissage dans le supérieur est incontestable

tous les cursus et les niveaux de diplômes les plus élevés. Pour autant, nous ne pouvons ignorer certaines dérives, en particulier la manière dont certains établissements privés lucratifs captent massivement les aides à l’apprentissage. Ces structures, parfois très éloignées des standards de qualité et d’accompagnement attendus, bénéficient des mêmes niveaux de soutien public que les CFA des chambres consulaires ou les établissements publics. Nous saluons la volonté du Gouvernement de réformer le modèle de financement, en limitant les excès, en encadrant les marges, en rétablissant l’équité entre les acteurs. Il faut assurer une juste allocation de l’argent public, au service de l’intérêt général et non au bénéfice de stratégies commerciales. L’apprentissage doit aussi être un levier de développement local. la Loire Atlantique compte des filières clés : l’industrie navale, l’agroalimentaire, le bois, l’économie circulaire ou l’économie du soin. Ces secteurs appellent à l’ouverture de nouvelles formations, construites avec les entreprises, les branches, les chambres consulaires et les collectivités. Dans certains territoires, il existe aussi des besoins de formation spécifiques, dans des secteurs de niche. Leur développement et la transmission des savoirs pourraient être mieux accompagnés grâce à des filières d’apprentissage. Je pense ainsi au métier

concernera les seuls contrats en cours. Ces changements alignent le régime des apprentis sur celui des stagiaires. Ce choix politique injuste pèse sur la dynamique de l’apprentissage, notamment dans les secteurs les plus fragiles, comme l’artisanat, où chaque euro compte dans la décision de recruter ou non un apprenti. faire preuve d’une vigilance accrue sur la mise en œuvre de cette réforme, pour qu’elle ne vienne ni freiner l’essor de l’apprentissage ni décourager les entreprises, qui, au quotidien, forment et accompagnent la jeunesse de notre pays.

son rôle de transmission est reconnu. Il est aussi tourné vers l’innovation. Il faut valoriser celles et ceux qui choisissent l’apprentissage, mais aussi tous ceux qui s’engagent pour que cette modalité de formation soit de grande qualité et à la portée de tous, qu’ils soient formateurs ou maîtres d’apprentissage. Nous devons continuer à promouvoir une vision exigeante et humaniste de l’apprentissage : ancré dans les territoires, ouvert à tous, équitablement financé et au service du bien commun. je vous remercie

catégories socio professionnelles les moins qualifiées, mais il ne faut pas décourager l’embauche d’apprentis au plus haut niveau de qualification, ces derniers méritant aussi une reconnaissance de leur diplôme et de leur engagement dans ce type de formation.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, qui, dans cet hémicycle, a conseillé ou conseillerait à ses enfants de choisir un lycée professionnel ou un CFA plutôt qu’un lycée général ou une grande école ?

Maintenant, gamin, ce n’est plus possible : plus tu feras d’études, moins tu bosseras et plus tu gagneras. » Qui n’a jamais entendu ces paroles ? En 2018, on a choisi de réformer l’apprentissage pour en faire une voie d’excellence, un moyen de lutte contre le chômage des jeunes et une politique d’émancipation sociale.

est donc important de passer par l’apprentissage. Mes chers collègues, vous l’avez compris, je lance un cri du cœur, car j’en ai assez que l’on dévalorise la voie professionnelle et l’apprentissage. Si ce dénigrement est malheureusement parfois sincère, il est souvent l’expression d’une forme de résignation plus profonde, directement liée à la réalité de notre culture de l’entreprise et de l’entrepreneuriat. L’apprentissage, c’est un trampoline : il peut vous faire décoller très rapidement et, dans tous les cas, vous retomberez sur vos pieds.

devrait être une fusée vers l’entrepreneuriat et les postes à responsabilités. Aujourd’hui, vous voulez monter votre boîte après avoir roulé votre bosse dans une TPE PME – je pense au bâtiment bien sûr, mais pas seulement – ? Eh bien, vous vous cognez les délais de l’administration,

Vous voulez intégrer une grande boîte par la technique et monter en compétence ensuite ? Ce n’est plus possible – en tout cas, c’est devenu trop rare. On vous répondra que l’on préfère embaucher un ingénieur ou un bac+5 pour faire votre boulot plutôt que de vous faire monter en interne.

J’entends souvent que les jeunes n’ont plus le goût de l’effort. Comment leur donner tort quand, dans notre pays, le système est tel que l’on préfère passer plus de temps à éviter de perdre de l’argent plutôt qu’à en gagner, à chercher les niches fiscales plutôt qu’à produire de la richesse ? C’est vrai ! À la fin, c’est notre pays qui tombe en ruines. Ce n’est pas aux jeunes de changer ; c’est à nous de revoir notre logiciel, notre façon de penser et de faire, pour valoriser le goût de l’effort, du risque et de la réussite.

La commission des affaires sociales a fait siennes nos conclusions. Nous y avons notamment pointé la réforme de 2018, qui, certes, a amorcé une dynamique considérable en faveur de l’apprentissage, mais n’a pas anticipé ses besoins de financement.

nous en sommes tous persuadés : il faut encore et toujours encourager l’apprentissage. La supériorité d’un enseignement par la pratique est d’autant plus manifeste qu’elle s’adresse à tous les publics, notamment ceux qui peuvent se trouver en difficulté.

Pour ce faire, madame la ministre, je propose depuis longtemps et de manière constante plusieurs solutions qui se déclinent dans le temps. Premièrement, il convient de ne donner à France Compétences que deux missions claires : l’apprentissage et le CPF.

de stopper cette logique de guichet en arrêtant les compteurs au financement de 900 000 apprentis, tout en considérant que le CPF a trouvé son rythme de croissance. Cette logique permettra de désendetter France Compétences et de cesser les changements permanents de financements, notamment sur les coûts contrats, rendant aujourd’hui fragile, complexe et parfois illisible le financement de l’apprentissage.

ensuite, la relance d’une concertation entre les régions, les CFA, les organisations professionnelles et les organisations syndicales, aux fins de trouver des marges de manœuvre supplémentaires

Mme la ministre.

pour l’avenir professionnel de nos jeunes, en particulier dans un contexte où leur insertion sur le marché du travail constitue un défi majeur. Elle est est aujourd’hui un levier essentiel d’insertion sociale et professionnelle. Poursuivons les efforts engagés pour développer cette voie, qui attire de plus en plus de jeunes gens dans notre pays. l’apprentissage en France a connu une progression significative ces dernières années, permise par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et par le dispositif « 1 jeune, 1 solution près de 880 000 contrats ont ainsi été signés, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à 2023. Ce chiffre témoigne du succès du modèle.

Un décret publié le 23 février dernier fait évoluer les aides à l’embauche. Celles ci passent de 6 000 euros à 5 000 euros pour les petites entreprises et à 2 000 euros pour celles de plus de 250 salariés. décret, publié voilà seulement quelques jours, modifie quant à lui le système d’exonérations de cotisations sociales salariales, en application de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale

alors que le signal envoyé au monde économique ne vienne briser la bonne dynamique de l’apprentissage. L’enjeu est clair : il faut trouver un équilibre entre la nécessaire maîtrise des finances publiques et le maintien d’un niveau d’apprentissage élevé élevé au service de l’emploi des jeunes et de la compétitivité de nos entreprises. Une évolution des politiques de soutien à l’apprentissage est elle pour autant malvenue ? Non, de toute évidence. Au delà des aides, il est essentiel de continuer d’investir dans la qualité des parcours, dans l’orientation et l’accompagnement des jeunes, afin de garantir une insertion durable. Pour préparer cette intervention, j’ai rencontré la semaine dernière la présidente et le directeur du centre de formation des apprentis interconsulaire de l’Eure de Val de Reuil. Véritable modèle de réussite, cet établissement est l’un des plus grands CFA de France. Nos échanges ont été riches. riches. L’abaissement du niveau des aides à l’embauche ne devrait pas dissuader les artisans et les petites entreprises de recruter des apprentis, en particulier dans les secteurs en tension.

Et si la hausse prévue des cotisations sociales a pour mérite de rationaliser les niveaux de rémunération, la question du financement de l’apprentissage demeure centrale. Madame la ministre, nous saluons à cet égard le bon déroulement des concertations que vous menez depuis l’automne dernier et qui devraient aboutir à la fin du mois d’avril. Leurs conclusions sont attendues par toutes les parties prenantes.

Dans le contexte budgétaire actuel, nous devons absolument orienter nos discussions vers un meilleur fléchage de ces dépenses, tout en préservant l’excellence du modèle français de l’apprentissage. J’emploie à dessein le terme d’excellence, car c’est le seul qui peut qualifier la voie de l’apprentissage dans notre pays. En conclusion, l’apprentissage reste un pilier central de notre politique de formation et d’emploi. Les ajustements à venir devront être pensés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs concernés pour continuer de faire de l’apprentissage un modèle satisfaisant pour tous. La parole

contestables ou discutables. L’apprentissage permet de former nos jeunes et de renforcer l’adéquation entre les besoins en ressources humaines des entreprises et les formations proposées.

Cet engouement s’explique par des politiques publiques particulièrement généreuses, qui se sont révélées être parfois en décalage avec les coûts réels de certaines formations du tertiaire ou les besoins en ressources humaines. Comme le constate la Cour des comptes, le cadre législatif a été rénové sans stratégie nationale ni financement adapté. L’objectif apparemment louable du Gouvernement d’atteindre le million d’apprentis n’a été associé à aucun critère d’utilité de la dépense.

Finalement, les 16 milliards d’euros que coûte annuellement l’alternance représentent un poids trop important pour France Compétences. Le déficit de cet organisme a justifié des baisses de prise en charge du coût des formations de façon quasiment indiscriminée.

des jeunes à l’emploi et contribuant à maintenir une économie dynamique dans les territoires. Nos jeunes artisans devront reprendre, dans les dix prochaines années, environ 300 000 entreprises, toutes importantes pour notre vie locale. Sans sauvegarde de notre modèle d’apprentissage, ce sont nos boulangers, nos cuisiniers, nos mécaniciens, nos charpentiers, nos plombiers, nos agriculteurs, et tant d’autres métiers encore, que nous pourrions voir disparaître de nos territoires.

Mme la ministre.

l’apprentissage est un levier puissant d’insertion et de réussite qui a fait ses preuves. Pour qu’il poursuive sa dynamique, encore faut il lever les freins que rencontrent les acteurs sur le terrain.

vers l’apprentissage. Pour certains jeunes, cette marche est bien trop haute. Nous avons donc là un levier à actionner. Alors qu’un jeune peut désormais passer son permis dès 17 ans, il doit attendre d’avoir 18 ans pour accéder à l’aide au financement du permis B. Cette incohérence pénalise particulièrement les jeunes issus des territoires ruraux, où la mobilité conditionne l’accès à la formation et à l’emploi.

qu’à apposer leurs signatures. Cette simplicité apparente peut masquer un déséquilibre. Un jeune en difficulté, parfois en position de fragilité,

Afin de mieux encadrer ces situations et d’assurer une médiation, prévoyez vous, madame la ministre, d’impliquer systématiquement les organismes de formation dans la procédure de rupture ?

de signer de nouveaux contrats, les aides aux entreprises étaient bloquées et les formations proposées ne figuraient plus sur la plateforme Parcoursup. Afin d’éviter que ces retards ne pénalisent des structures pourtant conformes et engagées, il pourrait être envisagé d’instaurer un délai de grâce de deux mois, dès lors que l’audit de renouvellement a bien été réalisé à temps. Cette mesure irait d’ailleurs dans le sens de la simplification administrative voulue par le Gouvernement, le Sénat et son président.

Les collectivités font face à des arbitrages douloureux. Elles auront le choix entre renoncer à l’apprentissage et… renoncer à l’apprentissage. Il est impératif de construire un modèle pérenne de financement à la hauteur des enjeux,

Mme la ministre.

448 000 à près d’un million. Cette réussite collective, fruit de la mobilisation des services de l’État, des régions, des CFA et du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat, contribue à redonner à l’apprentissage C’est heureux, car, outre une formation diplômante et une rémunération, cette voie de formation assure une insertion rapide et durable dans le monde du travail.

De fait, des milliers de jeunes accèdent à de hauts niveaux de qualification et à des formations d’excellence alors qu’ils n’en auraient pas eu les moyens autrement. Toutefois, cette ambition a un coût faramineux : 25 milliards d’euros en 2024 selon certaines estimations.

exigences quant à la qualité des formations dispensées en alternance. Le développement rapide de l’offre, facilité par une certaine forme de dérégulation – disons les choses –, se caractérise par l’émergence d’une multitude d’établissements d’enseignement à but lucratif, dont certains n’ont d’autre objectif que le rendement financier. Certaines structures tirent profit de cet effet d’aubaine, en l’absence de véritable contrôle de la qualité pédagogique. Dans un rapport d’information de 2024, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a ainsi déploré un « contrôle qualité défaillant » et un niveau de prise en charge identique pour les formations rigoureusement encadrées et pour celles dont les standards pédagogiques sont discutables. Il est donc impératif que l’optimisation du soutien public à l’apprentissage repose sur des critères objectifs liés à la qualité réelle des formations, à l’encadrement pédagogique, à l’agrément des établissements et à l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des diplômés. C’est dans cet esprit que j’ai fait adopter un amendement à la loi de finances pour 2025 visant à réduire le niveau de prise en charge des formations dispensées intégralement à distance. La France doit continuer de nourrir une ambition forte en matière d’apprentissage. Ce dernier doit être non pas un marché, mais bien une voie royale d’accès à l’emploi et un vivier de compétences pour nos TPE,

de certifier les établissements privés respectant des critères exigeants. Le Gouvernement semble avoir récemment renoncé à cette idée, au profit d’un renforcement de l’agrément Qualiopi. Or les limites de Qualiopi sont connues : lourdeur administrative, coût élevé, fraudes, prolifération d’organismes de certification peu scrupuleux. Dès lors, madame la ministre, comment garantir que les fonds publics alloués à l’apprentissage bénéficient aux établissements réellement engagés dans la réussite des jeunes, et non à ceux qui ne poursuivent qu’une logique de profit à court terme ? Par ailleurs, pouvez vous nous éclairer sur la manière dont vous entendez renforcer le dispositif Qualiopi ?

Chacun se souvient du dilemme cornélien auquel nous faisions face il y a quelques mois, lors de nos débats budgétaires ô combien difficiles, au sujet d’une politique fondamentale : la formation professionnelle des jeunes. réduire les dépenses de l’État en sabrant les aides en faveur de l’apprentissage ou maintenir ces aides sans contribuer à l’effort de réduction des dépenses ? Au cours cours des auditions réalisées par la délégation sénatoriale aux entreprises et la commission des affaires sociales, nous avons unanimement constaté le bénéfice de l’apprentissage. Sa remise en cause totale aurait été désastreuse. j’avais déposé des amendements visant à moduler le montant des aides suivant la taille des entreprises. Madame la ministre, vous avez été à l’écoute de mes propositions et vous avez tenu vos engagements. En effet, le Gouvernement a décidé de reconduire par décret l’aide aux entreprises qui emploient des apprentis selon un barème juste et proportionné : cette aide s’élève à 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés, à 2 000 euros pour les autres entreprises, à 6 000 euros pour toutes les entreprises accueillant un apprenti en situation de handicap. apprenti en situation de handicap. Par ailleurs, un décret publié le 28 mars dernier prévoit l’exonération de la totalité des cotisations salariales pour les rémunérations inférieures ou égales à 50 % du Smic, contre 79 % auparavant.

Aujourd’hui, plus que jamais, dans un monde en plein chahut, nous avons conscience que l’avenir est source de préoccupations, quels que soient votre niveau de diplôme et le secteur d’activité dans lequel vous évoluez. Vous êtes l’avenir de notre nation et notre priorité accompagner. Madame la ministre, nous devons être vigilants sur la qualité de l’apprentissage, parce qu’il s’agit de mobiliser de l’argent public et surtout parce qu’il y va de l’avenir de la jeunesse. Être attentif à la qualité des enseignements, c’est ne pas laisser la place à des structures peu scrupuleuses qui profiteraient du système sans être à la hauteur des enjeux. Comment les opérateurs de compétences et l’État peuvent ils mieux contrôler, et plus fermement, les organismes de formation privés qui accompagnent des apprentis ?

Nous devons éviter le raccourci selon lequel les petites entreprises embaucheraient des apprentis à de petits niveaux de diplômes. Leur besoin d’apprentis ayant un haut niveau de qualification est bien réel. Ne nous méprenons pas

Mme la ministre. Monsieur le président, madame

trop d’entreprises peinent aujourd’hui à recruter. Trop de jeunes doutent de leur avenir et, il faut le dire, dans la France de 2025, trop de déterminismes sociaux pèsent encore sur notre système éducatif. Trop de talents passent entre les mailles du filet simplement parce que l’on n’a pas su les orienter ni les former. Le premier pas dans le monde du travail est souvent celui qui lance un jeune dans la vie d’adulte. Le travail – faut il le rappeler ? – nous responsabilise, nous émancipe

de chômage des jeunes de 15 à 25 ans s’élevait encore à 19 % au quatrième trimestre de 2024, un taux deux fois supérieur à la moyenne nationale. Nous devons aujourd’hui relever les défis spécifiques auxquels les jeunes font face sur le marché du travail, comme l’a souligné ma collègue Marie Do Aeschlimann. Cela suppose de réconcilier l’école et l’entreprise. Nous devons briser un tabou, en instaurant une coopération accrue entre les acteurs de l’éducation, de la formation professionnelle et du monde économique. L’enjeu consiste d’abord à valoriser l’apprentissage, plus tôt et auprès du plus grand nombre. L’apprentissage n’est pas une voie de garage ni une simple alternative à la voie universitaire. C’est un chemin concret vers l’emploi, l’acquisition de savoir faire et l’indépendance. Il progresse d’ailleurs dans tous les secteurs, que ce soit dans l’artisanat, le tourisme ou les services. Développer l’apprentissage, c’est rendre plus accessible la première embauche, c’est aussi relancer l’emploi. C’est permettre la transmission des petites entreprises et le développement des plus grandes.

pour les apprentis qui a été décidée lors de l’examen du budget. Si ces ajustements fiscaux visent à optimiser les dépenses publiques, ils doivent demeurer un soutien à l’apprentissage et un levier clé pour l’insertion professionnelle des jeunes. N’oublions pas que l’embauche d’un apprenti constitue un investissement non négligeable, notamment pour les entreprises de moins de 250 salariés, qui emploient aujourd’hui près de 80 % des apprentis. À Paris, la ville doit pouvoir prendre toute sa part à cette dynamique. Je pense notamment à la création de partenariats avec des CFA pour adapter l’offre de formation aux besoins économiques de la capitale. L’enjeu est également de favoriser l’apprentissage dès l’enseignement secondaire. Nous devons réfléchir à la création d’un statut scolaire de l’apprentissage. Ce dernier devrait être possible dès l’âge de 14 ans, sans condition, pour mieux orienter les collégiens vers une filière en lien avec leurs compétences. Enfin, en matière de pilotage des politiques liées

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le président de la commission de la culture, de l’éducation et des sports, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur

que nous sommes parvenus au terme de ce débat, je tiens à vous remercier pour la précision de vos questions, qui prouvent combien votre assemblée est engagée et exigeante sur ce sujet. Je salue la ténacité du président Larcher qui a réussi à relancer les Rencontres sénatoriales de l’apprentissage, qui n’avaient plus eu lieu depuis la crise sanitaire. Ce débat dans l’hémicycle nous a permis d’aller au fond des choses, davantage que lors des discussions budgétaires, Depuis 2018, nous avons lancé une révolution de l’apprentissage en adaptant les dispositifs en place, en amplifiant le soutien budgétaire et en changeant surtout les mentalités. Désormais, nous devons consolider les acquis de cette révolution, dans un contexte qui exige un sens aigu de la responsabilité budgétaire. Après une phase d’extension et d’expansion de l’apprentissage, nous devons aujourd’hui améliorer le dispositif sur plusieurs points clés : l’adéquation

doit être évalué au regard des besoins des entreprises, des artisans et de notre pays. Beaucoup de professions, certaines filières parfois, connaissent des tensions de recrutement. Pour réaliser les quatre transitions que nous traversons – démographique, numérique, écologique et stratégique –, dans le contexte géopolitique que nous connaissons,

La remise à plat de la certification Qualiopi, en lien avec le ministère de l’enseignement supérieur, nous permettra, grâce à de meilleurs indicateurs, de mieux garantir que les formations répondent aux besoins des entreprises et aux attentes des apprentis et facilitent l’insertion professionnelle

de six mois, les perspectives d’insertion professionnelle dans un emploi, les rémunérations attendues et les différents métiers proposés. Le pilotage par la qualité, qui permet la meilleure adéquation entre l’offre et les besoins, implique de renforcer le rôle des entreprises et des

communiquer dans un cadre juridique sécurisé sur les contrôles qu’ils réalisent. La réactivité et la coordination des actions sont absolument centrales pour lutter efficacement contre les organismes fraudeurs.

la nécessité de porter un « autre regard » reste d’actualité. Il est important de travailler sur l’image que renvoient l’apprentissage et les métiers de l’artisanat. Même si l’on constate une légère amélioration, les métiers manuels restent, dans notre système scolaire, mal appréciés, car souvent mal connus. Plus généralement, cette situation pose la question de la découverte des métiers et de l’orientation des jeunes. Pour un trop grand nombre d’entre eux, l’orientation reste subie et non pas choisie. Par ailleurs, si l’apprentissage présente un bon taux d’insertion professionnelle, il reste un modèle fragile, qui a besoin de prévisibilité. Selon les chiffres de la Dares, les entrées en apprentissage ont baissé de 14 % en janvier 2025. Les nombreuses hésitations d’ordre budgétaire, lors de l’examen du projet de loi de finances, que ce soit sur le le montant de l’aide allouée, la taille des entreprises concernées ou le niveau de diplômes des jeunes, ont secoué le monde de l’apprentissage. Dans ces conditions, chacun ici comprend la position attentiste

de l’état des finances publiques et du coût de la politique de l’apprentissage. Aussi, au nom de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, je réitère nos mises en garde concernant l’enseignement supérieur privé lucratif,

séance par l’examen, sous la présidence de M. Pierre Ouzoulias, des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire.

Monsieur le président,